qui siégea au sein du groupe de l’Union centriste des démocrates de progrès, puis de l’Union Centriste, et qui fut questeur du Sénat. Ce médecin de formation, professeur agrégé à la faculté de médecine de Nancy, était un grand humaniste. Pionnier, il s’impliqua dans des sujets qui demeurent d’actualité : la lutte contre le cancer, les greffes ou encore les questions de bioéthique. Il créa ainsi le centre d’hémodialyse de Nancy, où il réalisa les premières transplantations rénales. Il présida l’Institut Curie jusqu’en 2013 et siégea notamment au Comité international de bioéthique de l’Unesco entre 2002 et 2006. Au Sénat, il s’investit tout naturellement dans les questions de santé et de bioéthique au sein de la commission des affaires sociales, dont il fut le vice président.

Au nom du Sénat tout entier, je veux assurer sa famille et ses proches, ainsi que le président et les membres du groupe Union Centriste, de notre sympathie. C’est aussi avec une grande tristesse que nous avons appris le 12 octobre dernier le décès de notre ancien collègue Jean François Picheral, qui fut sénateur des Bouches du Rhône jusqu’en 2008. Médecin radiologue de profession, il siégea au conseil général des Bouches du Rhône et fut élu maire d’Aix en Provence en 1989. Durant ses deux mandats de maire, Jean François Picheral a contribué au lancement de projets structurants pour sa ville, comme la requalification du cours Mirabeau ou encore l’implantation de la gare TGV sur le plateau de l’Arbois. Élu sénateur en 1998, Jean François Picheral fut secrétaire de la commission des affaires culturelles et vice président de l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé.

aux légionnaires, de devenir français de plein droit, s’il le souhaite, sur proposition du ministre de la défense. Il voyait dans le service sous nos drapeaux une preuve incontestable de l’attachement porté à notre pays

chaque 13 juillet, dans le jardin du Luxembourg. Au nom du Sénat, je salue la mémoire d’un homme engagé pour son territoire et ses habitants, et j’adresse mes condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches. En ces semaines

C’est sans doute une première dans l’histoire du Sénat, mais l’actualité et la menace sans précédent qui pèse sur les agriculteurs français la justifient

au beau milieu des manifestations agricoles et avant les élections européennes, c’est lui qui assurait que les négociations avec le Mercosur étaient suspendues. C’est encore lui qui s’engageait à ce que cet accord ne soit pas conclu sans clauses miroirs, ces dispositions dont on parle tant, mais qui n’existent toujours pas.

Comme l’a confirmé dans la presse Mme la ministre Primas le 22 octobre dernier, les textes sont clairs : les accords d’association comme celui qui a été négocié avec le Mercosur sont des accords mixtes, qui nécessitent une approbation à l’unanimité des États membres au Conseil de l’Union européenne. ! Si nous savons bien que la Commission européenne entend contourner ce veto en scindant l’accord pour isoler son volet commercial, aucune décision officielle n’a été prise à ce jour.

Pourquoi n’exercez vous pas le veto qui vous revient de plein droit ? Il faut conclure ! Enfin, combien de temps encore allez vous nous contraindre, nous, représentants élus du peuple français, à regarder périr nos agriculteurs et nos entreprises, en acceptant que cette Commission européenne outrepasse ses droits et piétine la démocratie ?

Un blackout total de près de quarante huit heures, provoqué par l’arrêt brutal des moteurs de la centrale EDF PEI de la Pointe Jarry, a laissé 230 000 foyers et leurs habitants sans électricité ni lumière, livrés à eux mêmes dans une nuit interminable. Dans cet instant suspendu, nos concitoyens ont vécu la peur, l’angoisse et l’insécurité. Des pillages, des saccages et des actes de vandalisme se sont multipliés dans les rues de Pointe à Pitre, malgré le couvre feu décrété par le préfet de Guadeloupe. Certains sont allés, impunément, jusqu’à utiliser une pelle mécanique pour détruire une bijouterie en plein centre ville. Imaginez, monsieur le ministre, des familles, des enfants terrifiés, des malades en détresse dans des hôpitaux fonctionnant grâce à des générateurs d’urgence à l’autonomie incertaine. Cette situation chaotique a cruellement exposé des failles dans la sécurisation de nos sites stratégiques et la vulnérabilité de nos territoires face aux tensions sociales et aux crises énergétiques. Ce drame interroge comment, en 2024, des citoyens peuvent ils être ainsi abandonnés, sans défense, dans le noir et l’impuissance ? Je condamne sans concession ces actes de sabotage. Aucune revendication ne saurait légitimer de telles actions, quels que soient les griefs des parties. Il est impératif de retrouver le chemin du dialogue et d’entamer des négociations respectueuses de l’intérêt général. Aussi, monsieur le ministre, ma question est simple : quelles mesures seront prises pour garantir que de telles structures d’intérêt public ne soient plus jamais menacées et que de tels événements ne puissent plus se reproduire ?

des infrastructures ferroviaires et routières, mais aussi de leur adaptation au changement climatique. À la demande du Premier ministre et de la ministre Catherine Vautrin, j’organiserai, au début de l’année prochaine, une conférence sur le financement des mobilités. Celle ci permettra, je l’espère, de mettre davantage en adéquation

de la route, en mettant plus de personnes dans moins de véhicules. C’est tout l’enjeu du plan Cars express, que j’ai l’intention de présenter au début de l’année 2025 et qui doit mobiliser l’ensemble des collectivités locales aux côtés de l’État. J’espère que les débats qui se dérouleront dans les assemblées à l’automne déboucheront

et Social Européen. Madame la ministre, le plan Marseille en grand, estimé à 5 milliards d’euros et lancé en septembre 2021 par le Président de la République, apportait une réponse forte de l’État à des carences anciennes, ainsi qu’à des retards importants dans le développement des services structurants pour la population de l’agglomération marseillaise : écoles, transports, logement ou encore sécurité.

J’alerte simplement sur les défis que pose un tel plan. Marseille, ville que l’on aime ou que l’on déteste, est une porte d’entrée de l’Europe depuis la Méditerranée. Ce positionnement stratégique nous impose une obligation de résultat dans l’exécution d’un plan dont la Cour des comptes elle même souligne le caractère indispensable. Ne gâchons donc pas notre chance de voir la deuxième ville de France se redresser. La renaissance de cette cité profitera à tous et rejaillira sur l’ensemble des communes du département, sur la région et sur la France. Aussi, madame la ministre, ma question est simple : suivrez vous la préconisation judicieuse de la Cour des comptes relative à la création d’une superstructure de gouvernance accompagner, malgré les temps difficiles, le versement des 5 milliards d’euros promis par le Président de la République ? La parole est à Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Madame la sénatrice

Mireille Jouve, pour la réplique. Madame la ministre, la sacralisation des financements et une superstructure de gouvernance : voilà ce qu’attendent les communes des Bouches du Rhône, qui n’ont pas les reins assez

et Républicain. Monsieur Guillaume Kasbarian, vous êtes ministre de la fonction publique et de l’action publique. On pourrait donc imaginer que votre priorité soit le service public, son efficacité, son excellence et son déploiement dans tous les territoires.

On pourrait imaginer que votre souci soit que les policiers ne se suicident plus et que les magistrats ne meurent pas d’épuisement en pleine audience. On pourrait imaginer que votre ambition soit de redonner aux Français le goût d’entrer dans la fonction publique. On pourrait imaginer que votre exigence soit d’assurer aux fonctionnaires l’estime et le respect des usagers, ce qui leur assurerait la sécurité au travail. Or, depuis votre prise de fonction, vous n’avez que le mépris à la bouche ! Comme si notre société n’était déjà pas assez divisée À coups de sur les arrêts maladie et les prétendus privilèges, à coups de comparaisons mensongères entre les salariés du privé et ceux du public, vous essayez de faire porter sur les fonctionnaires la responsabilité de la dégradation des services publics que vous avez consciencieusement organisée depuis 2017, vous et les gouvernements successifs que vous avez soutenus. Aussi, ma question est simple, monsieur le ministre : êtes vous là pour détruire la fonction publique, l’offrir au privé et éteindre derrière vous les lumières de la République ?

madame la sénatrice, des mesures d’accompagnement en matière de conditions de vie au travail, d’ergonomie des postes et de lutte contre les risques psychosociaux. Ce plan, c’est aussi une lutte contre la bureaucratie, qui

prochain, afin de « laisser la place à une nouvelle génération », comme il me l’a lui même dit et écrit. Je le remercie de son engagement au sein du bureau du Sénat, en tant que secrétaire, et au sein de la commission des finances, dont il a été l’un des vice présidents et un membre reconnu et, je dois le dire, apprécié. Il a contribué à de très nombreux travaux du Sénat sur des sujets financiers et fiscaux, en particulier en tant que rapporteur de la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales. Je lui souhaite le meilleur pour la suite,

Interrogé par un journaliste sur la chute de la bourse en cette fin d’année 1966, le président eut cette formule devenue célèbre : « La politique de la France ne se fait pas à la corbeille.

Le lendemain, deuxième lame : « Budget 2025 : Michel Barnier se lance dans la bataille politique sous l’œil des marchés financiers. » Madame Laurence Garnier, vous êtes membre du Gouvernement, mais je vous pose cette question très simple : est ce bien vous qui gouvernez encore ?

tout en vous remerciant, au nom de l’ensemble du Gouvernement, de votre engagement au cours de vos treize années de mandat.

Cette situation ressemble furieusement à de la dette perpétuelle. Le poids des marchés sera encore supérieur l’année prochaine. La République est chez Cofidis ! Voilà des décennies que les gouvernements s’ingénient à désarmer fiscalement l’État. En supprimant des impôts, nous avons ainsi perdu des centaines de milliards d’euros, qui nous manquent aujourd’hui pour rééquilibrer le budget. Et voilà cinquante ans que cela dure ! Il est grand temps de redonner à la République sa souveraineté fiscale et budgétaire. La dette, c’est le revolver de la finance qui met en joue les populations. Mesdames, messieurs les ministres, je laisse à votre sagacité cette citation de John Adams, qui fut le deuxième président des États Unis : « Il y a deux manières de conquérir et d’asservir une nation : l’une est par les armes, l’autre est par la dette. »

La suite, nous la connaissons tous : dans la périphérie rennaise, à dix minutes de ma commune de Pleumeleuc, une course poursuite s’amorce, des coups de feu éclatent, les assaillants prennent la fuite. L’enfant est touché à deux reprises à la tête. Son pronostic vital est toujours engagé. Il s’agit, j’y insiste, d’un enfant de 5 ans… Nos pensées vont évidemment à sa famille. Cette fusillade marque un nouveau palier dans la violence et l’horreur suscitées par le narcotrafic. Les narcotrafiquants ont désormais un coup d’avance sur les responsables politiques, et cela en dépit du travail quotidien et exceptionnel des forces de l’ordre et de la justice, auxquelles il faut rendre hommage.

La guerre à mener est transpartisane ; nous devons la conduire tous ensemble. Sinon, l’image qui risque de s’imposer dans l’opinion est celle d’un pays jalonné par les faits divers liés au trafic de drogue, tant dans nos villes que dans nos campagnes.

Je veux aussi avoir une pensée pour sa famille, pour ses proches, pour ce territoire que vous connaissez bien. L’idée qu’un enfant de 5 ans

! Cette tragédie montre malheureusement combien le ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, a eu raison de dénoncer les ravages du narcobanditisme dans notre pays – j’irai même jusqu’à parler, dans ce cas précis, de narcobarbarie. Je veux redire notre détermination à engager tous les moyens dont nous disposons pour lutter contre ce fléau. À cet égard, la proposition de loi déposée par les sénateurs Blanc et Durain constitue une base de travail tout à fait intéressante.

Enfin, madame la sénatrice, si vous me le permettez, je veux rappeler, comme le ministre de l’intérieur l’a déjà fait, qu’il existe un lien entre la consommation de drogue et le développement de ces réseaux mafieux. Il faut le dire clairement : aujourd’hui, dans notre pays, acheter de la drogue, c’est armer les trafiquants de drogue. Voilà la réalité

Quatre jours auparavant, un jeune de 15 ans avait été tué par balle dans le centre ville de Grenoble. Au début du mois d’octobre, un corps calciné a été retrouvé à Marseille. Ces drames, liés au trafic de drogue, terrifient les habitants. Depuis les petites communes jusqu’aux métropoles, le trafic s’est généralisé, la violence qu’il suscite. Les habitants exigent la sécurité, et ils y ont droit. Si nous saluons l’action de la police pour protéger nos concitoyens et lutter contre le trafic, la stratégie actuelle est un échec.

montre que la coordination avec les élus locaux, loin des polémiques stériles, donne des résultats. Le ministre de l’intérieur leur doit de la transparence sur le nombre des policiers nationaux déployés,

ne s’opposent pas ; ils se complètent. Allez vous enfin aborder cette question dans sa globalité, être transparent sur votre action, donner des moyens aux collectivités et faire confiance aux acteurs de terrain ?

tout d’abord excuser l’absence du Premier ministre. J’ai l’honneur de le représenter devant vous aujourd’hui et de répondre en son nom.

comme au niveau européen, à l’échelle du pays comme à celle de nos territoires, ainsi que vous venez de le rappeler. De plus en plus de villes sont touchées, y compris dans la profondeur du pays, loin des zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires où cette criminalité prenait traditionnellement appui.

Le Gouvernement s’est saisi de la question dès sa prise de fonction. Celle ci constitue l’une des priorités assumées par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale, que j’ai eu l’occasion de lire en son nom devant vous. que garde des sceaux, c’est le premier chantier que je souhaite mener à bien, car, je le sais, un grand nombre de mesures concernent la justice. Celle ci doit avoir à sa disposition plus de leviers pour lutter efficacement contre ce fléau. Et il y a urgence.

étroit avec le ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, car les mesures à prendre concernent nos deux ministères. Nous devons agir en complémentarité, non en opposition. La réponse passera forcément par un renforcement des moyens de l’État. Il faudra associer étroitement les élus locaux, qui ont évidemment un rôle central à jouer pour que cette lutte multidimensionnelle soit efficace. Avec le ministre de l’intérieur, j’ai annoncé ici même, depuis ce banc, que nous nous rendrions ensemble

lors du Conseil européen qui s’est tenu il y a quelques jours, la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, a annoncé qu’une nouvelle directive Retour allait prochainement voir le jour.

ont reçu l’ordre de quitter le territoire des États membres de l’Union européenne. Pourtant, seuls 90 000 d’entre eux ont fait l’objet d’un éloignement effectif. Cela signifie donc que, l’année dernière, moins de 20 % des décisions d’expulsion ont été exécutées en Europe… Ces chiffres envoient naturellement un signal délétère. Ils confirment que poser le pied sur le sol européen, c’est quasiment recevoir l’assurance de pouvoir s’y maintenir, quand bien même une décision de justice ordonnerait le contraire. Ces chiffres renforcent chez nos concitoyens le sentiment que les États ont réellement perdu le contrôle de la situation. La politique de retour engage l’efficacité de l’ensemble de la politique migratoire, mais elle constitue l’un des

dans l’Union européenne doivent donc être vues, selon moi, comme un moyen pour aider notre pays à faire de nouveau respecter ses frontières, comme les actes de son administration et les décisions de sa justice. Monsieur le ministre, ma question est donc simple. Comment la France entend elle entrer dans ces nouvelles négociations et quelles seront ses lignes de force ? La parole

et l’ensemble de ses homologues européens, nous avons vu combien les lignes avaient bougé sur la nécessité de maîtriser les flux migratoires. Bien malin celui qui aurait pu distinguer les positions d’un ministre social démocrate de celles d’un ministre conservateur…

au détriment de la qualité du service aux patients. Notre système de santé publique s’effondre sous nos yeux : délais d’attente qui s’allongent pour les rendez vous, prises en charge tardives, trajets à rallonge, alors que les services de proximité ferment. Madame la ministre de la santé, vous êtes aussi chargée Le coup de rabot que vous assénez dans le PLFSS pour 2025 ne met il pas à mal le principe même de notre sécurité sociale, selon lequel chacun doit contribuer en fonction de ses moyens et bénéficier en fonction de ses besoins ? Et que répondez vous au cri d’alarme cri d’alarme des soignants et des patients, que nous relayons au nom des élus locaux et des citoyens

madame la ministre, tout ne va pas si bien ! Le service public de la santé a besoin de perspectives pour être

Le défi est colossal, mais il n’est pas seulement d’ordre financier si l’on veut parvenir aux fins que nous nous assignons : assurer le désendettement de notre pays sans obérer ni son attractivité ni sa croissance, et sans oublier les plus fragiles.

sur le territoire. Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je suis heureux de saluer en votre nom la présence dans notre tribune d’honneur d’une délégation du groupe d’amitié Allemagne France du Bundesrat,

La délégation est accompagnée par notre collègue Ronan Le Gleut, président du groupe interparlementaire d’amitié France Par leur dialogue régulier, le Sénat et le Bundesrat apportent une contribution importante à la relation entre la France et l’Allemagne, ainsi qu’au lien de nos deux pays avec la Pologne dans le cadre du triangle de Weimar des secondes chambres. Cette rencontre fait suite à la visite de la présidente du Bundesrat, Mme Manuela Schwesig, au mois de mai dernier. Nous nous sommes rendus ensemble aux célébrations du 79 anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, ainsi qu’au mémorial de la Shoah ; ce fut un moment particulièrement fort. J’ai moi même été invité à prendre la parole à Bonn devant le Président de la République fédérale et les ministres présidents des Länder. C’était le 7 septembre dernier, à l’occasion du 75 anniversaire du Bundesrat, dans l’enceinte où a été adoptée la Loi fondamentale allemande et où s’est tenue la première session de la Chambre haute. Ce moment de commémoration était également tourné vers l’avenir, pour réaffirmer notre ancrage européen commun et, plus que jamais, la pertinence du couple franco allemand. Pour prolonger cet élan, les commissions des affaires européennes de nos deux chambres ont tenu des réunions conjointes à Stuttgart et à Strasbourg. À l’agenda des discussions de cette rencontre, nos groupes d’amitié ont retenu plusieurs sujets d’actualité, dont les frontières et l’immigration, ou encore la coopération en matière d’intelligence artificielle – autant de défis d’intérêt commun. Nous réfléchissons par ailleurs au développement de nouveaux partenariats décentralisés innovants. Permettez moi, madame la présidente, chère Anke Rehlinger, de vous dire combien je me réjouis de nos rencontres à venir.

derniers vérifient que le danger est bien pris en compte par les plans de maîtrise sanitaire des exploitants, que des autocontrôles sont réalisés et que toutes les mesures de correction sont mises en œuvre lorsque l’on constate des taux supérieurs à la réglementation. Ensuite, se le problème de la réglementation. Il est important de rappeler que les teneurs maximales en mercure sont fixées par une réglementation à l’échelle européenne. Elles sont déterminées de manière à assurer

emploieraient plus de 450 000 personnes et coûteraient plus de 80 milliards d’euros en 2023, contre 50 milliards d’euros en 2012, soit une augmentation trois fois plus rapide que l’inflation, tout en excellant dans l’engraissement des cabinets d’études. y a un véritable engouement pour les agences ! Et cela vaut aussi pour les collectivités, friandes de GIP, de SEM ou d’agences de développement qui se concurrencent. « Réfléchir aux agences, c’est réfléchir à l’État », nous disaient les auteurs du rapport annuel du Conseil d’État en 2012. ans plus tard, réfléchir ne suffit plus. Au moins cinq agences sont chargées de l’agriculture et de l’alimentation. Dans le domaine de la biodiversité et de l’environnement, ces entités opèrent souvent indépendamment, mais sur les mêmes sujets.

sur l’effectivité de la simplification et de la transformation de l’action publique –, il est nécessaire, indispensable et urgent qu’un état des lieux soit réalisé, afin de rationaliser et de regrouper cette débauche de bonne volonté. À l’aune d’une stricte sobriété budgétaire et d’un énième projet de loi de simplification, nous avons bien entendu vos engagements et ceux du Premier ministre. Aussi, monsieur le ministre, quelle est votre capacité à faire bouger les lignes, et dans quel délai ? Lorsqu’il y a une volonté, il y a un chemin. Quel est le vôtre ?

Autant de raisons de redouter cet accord, qui pourrait être entériné dès novembre prochain. En France, ce traité suscite une opposition quasi unanime depuis 1999. Il menace notre économie agricole déjà fragile, notre souveraineté alimentaire et nos principes environnementaux. Sans réciprocité, sans clauses miroirs environnementales et sanitaires, les conséquences seraient désastreuses pour une agriculture française en détresse. Notre pays doit se faire entendre. Nos agriculteurs ne peuvent payer le prix de l’affaiblissement du Président de la République sur la scène internationale ! Un fonds d’indemnisation, sorte de cache misère, ne réglera rien. La France ne peut accepter les manigances de la Commission européenne, qui tente de scinder cet accord pour faciliter son adoption. Aussi, quelles mesures comptez vous prendre pour faire entendre la voix de la France ? Le Gouvernement usera t il de son droit de veto pour s’opposer à cet accord ? Comptez vous lancer le débat au Parlement comme le demandait mon collègue Jean Claude Tissot en janvier dernier, et dans quel délai ?

La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour le groupe Les Républicains. la vie associative. Des experts indépendants de l’ONU ont récemment considéré que l’interdiction du port du hijab dans les compétitions sportives en France était discriminatoire et devait être annulée. annulée. Outre que ces mêmes experts n’évoquent jamais l’emprise religieuse pouvant peser sur les jeunes femmes musulmanes qu’ils entendent protéger, une telle exigence va évidemment à l’encontre de nos principes républicains, en premier lieu la neutralité et la laïcité, de notre histoire ayant abouti à la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État. En juin dernier, votre prédécesseure, monsieur le ministre, rappelait que le port de signes ou de tenues à caractère religieux était proscrit pour les athlètes de l’équipe de France participant aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en cohérence avec la règle 50 de la Charte olympique. Un an plus tôt, le Conseil d’État avait jugé que les règlements des fédérations de football et de basket ball relatifs à la neutralité vestimentaire au niveau amateur étaient proportionnés et adaptés au contexte sportif. On le voit, un important édifice juridique a été bâti dans notre pays, mais une consolidation s’impose face à la multiplication des faits communautaires et des dérives séparatistes.

Monsieur le ministre, comptez vous réaffirmer les propos du Premier ministre, qui, dans son discours de politique générale, indiquait qu’il n’y aurait « aucun accommodement sur la défense de la laïcité » Et comment prévenir toute remise en cause de ce principe fondamental, y compris par des experts déconnectés des fondements de notre République ? La parole

qui se traduit par l’interdiction de manifester des convictions et opinions religieuses pour les agents de l’État, des collectivités et de toutes les personnes morales chargées d’une mission de service public. Le Conseil d’État, dont la jurisprudence fait évidemment foi dans notre pays, reconnaît que les fédérations sportives délégataires sont chargées d’une mission de service public et que, à ce titre, les équipes de France et les agents des fédérations participent à l’exécution du service public et sont donc soumis au principe de neutralité. Concernant les compétitions internationales, telles que les jeux Olympiques et Paralympiques, chaque fédération internationale est chargée de fixer les règles qui s’appliquent aux disciplines relevant de sa compétence. En France, s’agissant des membres des équipes nationales, nous restons attachés à l’application stricte du principe de neutralité.

manifestations. Certaines fédérations ont fait le choix, dans des conditions limitées et pour certaines compétitions, d’adopter des règlements limitant le port de signes politiques et religieux. S’agissant des autres licenciés, les règlements fédéraux de la Fédération française de basket ball et de la Fédération française de football sont conformes à notre cadre juridique. C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 29 juin 2024, dans laquelle il a confirmé qu’il était adapté et proportionné, pour les fédérations sportives, de prévoir, pour le bon déroulement des compétitions et manifestations qu’elles organisent ou autorisent, l’interdiction du port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. En l’état du droit, il revient donc aujourd’hui aux fédérations de déterminer au regard de leur situation spécifique les règles nécessaires pour faire primer les principes de la République sur toute autre considération. Je proposerai

d’extrême urgence sur le plan budgétaire. Madame la ministre, il arrive souvent que les lois environnementales ne prennent pas en compte la réalité du terrain. Or, pour limiter les dégâts et les risques pour les personnes, il faut faire plus en matière de prévention et d’anticipation du risque. Nous savons le faire, mais les contraintes législatives et normatives empêchent souvent la pleine réussite de ces projets. Ce qui vise à la survie de l’homme doit être priorisé. Voilà le cap qui devrait nous inspirer, nous, le législateur, et vous, le Gouvernement. Madame la ministre, sur quelle base avez vous fixé la somme de 75 millions d’euros ? Seriez vous prête à en augmenter le montant, si le coût des dégâts était finalement bien supérieur, comme on peut s’y attendre ? Envisageriez vous d’assouplir les règles d’accès au fonds Barnier, afin de répondre à la répétition des événements dans certains territoires ? Quelles Quelles mesures de simplification entendez vous mettre en place pour permettre aux élus locaux de faire davantage de prévention en matière de gestion des cours d’eau et des forêts, pour mettre enfin la protection des humains au centre des priorités ?

La séance est reprise. J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale aux entreprises a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement. la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes rassemblés cet après midi afin d’examiner la proposition de loi visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie, adoptée par l’Assemblée nationale le 16 avril 2024.

En France, le nombre de nouveaux cas de cancers détectés est estimé à 1 200 par jour sur une année. Un Français sur vingt est concerné, soit deux fois plus qu’il y a trente Les cancers représentent aujourd’hui la première cause de décès prématurés en France, la première cause chez l’homme et la deuxième chez la femme, les cancers les plus fréquents étant ceux de la prostate, du sein, du côlon rectum et du poumon. En France, une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie.

En 2021, 12 600 décès ont été enregistrés. Il s’agit de la première cause de décès par cancer, même si le nombre de décès a connu une baisse de 1,3 % par an entre 2011 et 2021. Dans la majorité des cas, le développement d’un cancer du sein prend plusieurs mois ; lorsqu’il est détecté tôt, il peut être guéri dans neuf cas sur dix et les séquelles peuvent être réduites. Trois programmes de dépistage organisé ont été mis en œuvre, avec des tests et des examens gratuits pour les cancers localisés. Ainsi, chaque année, 9 millions de dépistages des cancers sont réalisés en France. Le Gouvernement souhaite poursuivre dans ce sens, car dépister précocement, c’est

Vous le savez, certaines femmes présentent un risque plus élevé que d’autres de développer un cancer du sein, du fait d’antécédents familiaux ou personnels. Pour ces femmes, des modalités spécifiques de dépistage ont été définies par la Haute Autorité de santé (HAS), comme des mammographies à fréquence plus rapprochée. Ces mesures font partie des plans Cancer, pour lesquels l’État a mobilisé depuis 2004 des moyens considérables afin de réduire significativement le poids des cancers dans le quotidien des Français. La stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021 2030 a apporté de nouveaux moyens budgétaires. Cette stratégie fixe des objectifs inédits et évolutifs : diminuer de 60 000 par an le nombre de cancers évitables à l’horizon de 2040 réaliser 1 million de dépistages supplémentaires d’ici à 2025 ; réduire de deux tiers à un tiers la part des patientes souffrant de séquelles cinq ans après un diagnostic améliorer significativement le taux de survie des cancers de plus mauvais pronostic d’ici à 2030 ; mieux accompagner les conséquences des cancers et des traitements sur la qualité de vie des personnes en minimisant les séquelles. Et les résultats sont là : plus de trois quarts des actions prévues dans la feuille de route 2021 2025, financée à hauteur de 1,7 milliard d’euros, commencent à porter leurs fruits. Le cancer du sein est au cœur de cette stratégie. L’objectif est de favoriser une détection précoce et ainsi de mieux prendre en charge et d’augmenter les chances de guérison, d’améliorer l’efficacité et la rapidité du parcours de dépistage, grâce à la mise à niveau du parc de mammographes, tout en facilitant le développement d’outils innovants. De nombreuses actions de prévention sont aussi menées – elles sont particulièrement visibles en ce mois d’Octobre rose. Près de 20 000 cancers du sein pourraient être évités chaque année

Son adoption en l’état conduirait ainsi à rendre inapplicables le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur, la participation forfaitaire et les franchises sur les soins consécutifs à un cancer du sein ou à un parcours de soins global. entraînerait la mise en place d’un régime différencié pour une pathologie spécifique, ce qui remettrait en cause un principe fondamental, celui de l’équité de notre système de santé. L’exonération totale des frais de santé pour les patientes atteintes d’un cancer du sein pourrait entraîner une rupture d’égalité entre les patientes atteintes de cette pathologie et ceux qui souffrent d’autres maladies,

Je le rappelle, notre système actuel de prise en charge du cancer du sein vise d’ores et déjà à limiter le reste à charge pour les patientes. Le cancer du sein est reconnu comme une affection de longue durée. Ce statut permet une prise en charge à 100 % du ticket modérateur par l’assurance maladie pour tous les soins en lien avec cette ALD, selon le tarif de remboursement fixé par la sécurité sociale. Les patientes bénéficient également d’une dispense d’avance de frais, à l’exception des dépassements d’honoraires, qui peuvent être pris en charge par les complémentaires santé. Nous réaffirmons notre volonté de plafonner les dépassements d’honoraires pour toutes les consultations ou soins des patientes traitées pour un cancer du sein. Tel est l’objet de l’article 1 , que nous soutenons. De plus, deux mécanismes protecteurs existent aujourd’hui pour limiter les restes à charge des personnes en ALD devant s’acquitter des participations forfaitaires et des franchises : le plafonnement annuel à 50 euros et une exonération de ces frais pour les personnes les plus précaires, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S). Les organismes complémentaires peuvent prendre en charge, pour les assurés couverts par un contrat responsable, le forfait journalier hospitalier, qui s’élève à 20 euros par jour en hôpital ou en clinique et à 15 euros par jour dans le service de psychiatrie d’un établissement de santé, ce qui représente plus de 95 % des contrats.

sont actuellement menés. L’objectif est d’améliorer les spécifications techniques des produits et de permettre ainsi une meilleure qualité, un meilleur confort et de réduire le reste à charge. Enfin, un forfait de 180 euros permet de prendre en charge des bilans diététiques, fonctionnels, motivationnels ou encore des consultations psychologiques, dans le cadre du parcours de soins des patients traités pour un cancer.

En revanche, et le Gouvernement est engagé en ce sens, nous devons continuer de travailler à des solutions équitables pour tous les patients atteints de maladies graves.

Je vous remercie,

Cette pathologie figure parmi les plus coûteuses pour les assurées. De tous les cancers, il est celui qui expose le plus souvent à un reste à charge. Il s’agit en outre du cancer féminin le plus répandu : on estime qu’une femme sur huit sera touchée par cette maladie au cours de sa vie. En 2023, 700 000 femmes vivaient en France avec un cancer du sein, traité ou en traitement, ce nombre étant en constante augmentation. Si le vieillissement de la population en est l’un des premiers facteurs – 80 % des cancers se développent après 50 ans il faut également prendre en considération l’exposition accrue à des agents cancérogènes dans l’alimentation et l’environnement, qui pourraient expliquer notamment la forte incidence du cancer du sein dans les Antilles. Cet exemple démontre que les femmes ne sont pas égales face au risque du cancer et que leur exposition varie selon leur lieu de vie, mais également, et c’est un facteur particulièrement important, selon leurs conditions de travail. (Inserm) a ainsi récemment mis en lumière que le travail de nuit augmentait de 30 % le risque d’avoir un cancer du sein. Si certaines formes de cancers du sein, à l’instar des triples négatifs, sont associées à des pronostics plus plus défavorables, le taux de survie moyen atteint 90 % pour les cas pris en charge à temps. C’est l’occasion pour moi de rappeler l’importance déterminante du dépistage et de saluer la campagne Octobre rose,

On ne peut, je pense, rester insensible face au cancer du sein. Nous connaissons toutes et tous des proches, des membres de nos familles, des administrés, qui ont eu à affronter cette maladie et qui nous ont raconté les délais angoissants, les traitements éprouvants et, peut être, le reste à charge, qui est vécu, aux dires de certaines, comme une double peine. La proposition de loi que nous examinons ce jour, déposée par l’ancien député Fabien Roussel et adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale, a pour objet de renforcer la prise en charge des soins, des traitements et des frais liés à un cancer du sein. C’est un objectif louable, qui fédère par delà les clivages politiques. Je tiens à cet égard à saluer les discussions constructives que nous avons eues en commission et qui témoignent de notre préoccupation sincère et partagée. Pour répondre à la question du reste à charge lié à un cancer du sein, il convient d’abord d’en comprendre les causes. Les assurées atteintes de cette maladie relèvent du régime des affections de longue durée, comme tous les patients atteints d’une tumeur maligne. Cela leur ouvre droit à une prise en charge renforcée grâce à une exonération du ticket modérateur sur tous les actes en lien avec le cancer du sein. La chimiothérapie, la radiothérapie, la mammectomie et même la reconstruction mammaire sont dès lors prises en charge à 100 % de la base de remboursement Toutefois, le régime des ALD n’évite pas tout reste à charge : la participation forfaitaire, la franchise médicale ou les forfaits en établissements de santé subsistent, par exemple, de même que le ticket modérateur pour des soins sans lien avec l’ALD. s’ajoutent les dépassements d’honoraires, notamment ceux qui sont pratiqués lors d’une chirurgie reconstructrice. Non remboursés par l’assurance maladie et souvent mal remboursés par les complémentaires santé, ils représentent le poste de reste à charge le plus important. Ils s’élèvent en moyenne à 1 391 euros et peuvent, dans certains cas, atteindre 10 000 euros et provoquer un renoncement financier aux soins.

Sur ma proposition, la commission des affaires sociales a renforcé la portée juridique de l’article 1. Dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, cet article prévoyait qu’une attention particulière devait être portée, lors des négociations conventionnelles, aux dépassements d’honoraires pratiqués dans le cadre du traitement d’une ALD, notamment d’un cancer du sein. Désormais, cet article prévoit que les dépassements d’honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à la prise en charge d’un cancer du sein peuvent être plafonnés dans le cadre des négociations conventionnelles.

permettra de réduire considérablement le plus gros poste de reste à charge des patientes ; je me félicite donc de cette avancée notable. Les assurées doivent également supporter le coût de soins et de prestations

son montant, de 180 euros, ne permet pas un suivi dans la durée. Un amendement du président Mouiller, soutenu par le Gouvernement, vise, d’une part, à ouvrir ce forfait aux patientes en traitement actif d’un cancer et, d’autre part, à créer un parcours spécifique au cancer du sein

coûteux, mais cruciaux pour la santé et le bien être des patientes. Ainsi, pour les accessoires, il faut compter 60 euros pour un mamelon en silicone, 70 euros pour chaque soutien gorge postopératoire et à peu près la même somme pour des soutiens gorge adaptés au port d’une prothèse mammaire amovible, ce montant devant bien sûr être pour disposer des rechanges nécessaires, le tout n’étant, à ce jour, pas remboursé. La demande de rapport formulée à l’article 1 a le mérite d’attirer notre attention sur ces coûts incompressibles. Je pourrais aussi longuement m’étendre sur la liste et le coût des soins de confort : crèmes relipidantes pour apaiser les effets secondaires de la chimiothérapie, patchs pour masser les cicatrices et strips pour les protéger, vernis pour prévenir la chute des ongles, autant de postes de dépenses qui n’ont rien de superflu ou de confortable. Croyez moi, toutes les assurées concernées préféreraient s’en passer. Dans ces conditions, l’article 1 de la proposition de loi vise à rendre inapplicables aux patientes traitées ou suivies pour un cancer du sein la plupart des postes de reste à charge : participation forfaitaire, franchise médicale, ticket modérateur et forfaits en établissements de santé. Il prévoit, en outre, une prise en charge intégrale de l’ensemble des soins et dispositifs prescrits dans le cadre d’un cancer du sein, ce qui comprend notamment les soins de support, les prothèses capillaires et le renouvellement des prothèses mammaires. Je le sais, certains sur ces travées estiment qu’en réservant aux seuls patients atteints d’un cancer du sein un régime de prise en charge favorable, incluant des dépenses pesant sur tous les assurés présentant une pathologie lourde, cet article contreviendrait au principe constitutionnel d’égalité. raison pour laquelle le président de la commission des affaires sociales a déposé un amendement visant à renforcer la prise en charge des seules dépenses propres au cancer du sein et à créer un forfait pour les soins et dispositifs non remboursables et spécifiques à cette pathologie. J’ai eu l’occasion de le dire, je n’estime pas que ce texte soit incompatible avec le principe d’égalité, puisque je pense que la nécessaire amélioration des conditions de prise en charge du cancer du sein aurait pu constituer un premier pas avant l’extension progressive du dispositif à d’autres pathologies. Pour autant, mes chers collègues, j’entends vos doutes. Notre seule boussole doit être l’intérêt des patientes, lequel passe par la sécurisation juridique du dispositif afin de nous assurer que les avancées prévues puissent effectivement entrer en vigueur. Les amendements du président Mouiller, s’ils limitent la portée du dispositif, sont loin de le vider de sa substance. Ils permettent même de fluidifier sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le remboursement des sous vêtements adaptés. Ces mesures répondent, je le crois, aux préoccupations et aux attentes des patientes. Alors que le reste à charge des assurées traitées ou suivies pour un cancer du sein atteint aujourd’hui un niveau insoutenable pour une majorité d’entre elles, cette proposition de loi et les amendements que j’ai évoqués des mesures aussi utiles que nécessaires pour alléger ce fardeau. Aucun patient ne devrait se retrouver en difficulté financière du fait de sa maladie ou, comme c’est trop souvent le cas pour les femmes atteintes d’un cancer du sein, avoir à renoncer à des modalités thérapeutiques pour des raisons financières. C’est là, me semble t il, l’essence même du droit constitutionnel à la santé, issu du préambule de la Constitution de 1946. En ce mois d’Octobre rose, montrons que le Sénat peut, dans un esprit transpartisan qui l’honorerait, répondre présent pour renforcer la protection et la prise en charge des malades du cancer du sein. Dans la suite

Ce régime donne droit à une exonération du ticket modérateur, c’est à dire à une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale des actes en rapport avec Les chimiothérapies, radiothérapies et mastectomies sont ainsi intégralement prises en charge dans la limite des bases de remboursement, tout comme la chirurgie reconstructrice et la pose d’implants ou, dans certains cas, l’achat de la plupart des prothèses externes. Le reste à charge demeure néanmoins très important. Il est estimé entre 1 300 et 2 500 euros en moyenne par la Ligue contre le cancer. Il touche plus des trois quarts des patientes, soit davantage que tout autre type de cancer. Cela s’explique par différents facteurs, à commencer par les dépassements d’honoraires liés à des opérations de reconstruction mammaire ou à l’achat de certains dispositifs médicaux comme les perruques. Ces dépenses ne sont pas un luxe, elles répondent à un besoin vital : pour les femmes atteintes du cancer, c’est le moyen de ne plus porter dans leur chair les stigmates de la maladie en restaurant l’image qu’elles ont d’elles mêmes. Le reste à charge élevé est source de dilemmes pour de nombreuses malades. Certaines doivent faire des choix douloureux : près de 15 % des patientes qui renoncent à une reconstruction mammaire le font pour des raisons financières d’autres renoncent aux prothèses capillaires, dont la prise en charge – pour celles qui sont jugées convaincantes – repose en grande partie sur les complémentaires santé. Il faut ajouter à cela qu’une ALD est souvent synonyme de baisse des revenus. Beaucoup de malades basculent dans la pauvreté et une personne sur trois perd son emploi dans les deux ans qui suivent le diagnostic. Par ailleurs, n’oublions pas que le cancer du sein est aussi source de profondes inégalités territoriales. La vulnérabilité à la maladie est, par exemple, accrue dans les territoires ultramarins, en raison d’une offre de soins insuffisante, de diagnostics tardifs ou de difficultés de prise en charge. Ainsi, en Guadeloupe, la survie après cinq ans chez la femme est de 79 %, contre 88 % dans l’Hexagone, alors même que l’incidence de ce cancer demeure moins élevée. Pour nombre de patientes, recevoir des soins se fait au prix d’un séjour très coûteux en métropole. Je tiens personnellement à saluer les personnes et associations qui facilitent l’accueil de ces femmes. Ces inégalités s’étendent également aux facteurs de risque. En Guadeloupe comme en Martinique, il existe ainsi une forte suspicion de lien de causalité entre l’exposition au chlordécone et le cancer du sein. Je rappelle que ce lien a été établi pour le cancer de la prostate. L’adoption de ce texte changerait donc radicalement la vie des femmes atteintes en outre mer comme dans l’Hexagone. Sa version actuelle pose pose néanmoins plusieurs difficultés, notamment sur la question de la rupture d’égalité – nous avons été nombreux à le souligner. Nous soutiendrons donc l’amendement du président de la commission des affaires sociales à l’article 1, qui vise à vise à recentrer le dispositif proposé sur les frais spécifiques au cancer du sein, notamment ceux qui sont consécutifs à une mammectomie ou une tumorectomie. Nous soutiendrons également les amendements à l’article 1 qui tendent à inclure les patients en traitement actif pour un cancer dans le cadre du parcours de soins global et à déployer un parcours de soins spécifique et renforcé pour les assurés atteints d’un cancer du sein. Comme vient de le souligner Mme la ministre, un certain nombre de questions restent néanmoins en suspens, à commencer par la faisabilité technique et les potentiels effets de bord que ces mesures pourraient provoquer sur les autres ALD. Sous réserve de l’adoption des amendements du président Mouiller, le groupe RDPI votera ce texte à l’unanimité. Cette proposition de loi ne règle évidemment pas tout et pose des questions en matière d’égalité devant la maladie. Nous estimons qu’il faudra aller plus loin en se penchant sur l’ensemble des cancers et des autres ALD,

ce mois d’Octobre rose qui s’achève marque le vingtième anniversaire de la généralisation du dépistage organisé du cancer du sein. Cet anniversaire et cette proposition de loi sont l’occasion de rappeler que ledit dépistage sauve des vies, mais que son taux de réalisation n’atteint toujours pas 50 %, malgré les efforts de l’État et des collectivités

le plus meurtrier chez les femmes, l’un des plus mutilants aussi, et le plus répandu, ce qui justifie pour certains un traitement particulier, cette proposition de loi, en l’état, pose un vrai problème de rupture d’égalité. Comment expliquer à un patient atteint d’un autre cancer que sa prothèse capillaire ne sera pas prise en charge à 100 %, qu’il devra régler sa participation forfaitaire,

pour les patients atteints d’un cancer du sein, ce qui est une réelle avancée. Nous les voterons. L’activité physique adaptée étant mentionnée dans ces soins de support, j’en profite

Sophie Romagny. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en plein Octobre rose et alors que nous célébrons les 20 ans du dépistage généralisé du cancer du sein, nous nous exprimons sur la prise en charge des soins pour les patientes. Je remercie sincèrement notre rapporteure, Cathy Apourceau Poly, pour la qualité de ses travaux. Le coût de la maladie pour une femme est un aspect encore trop peu évoqué. Je viens vous parler, à mon tour, des 700 000 femmes qui, en 2023, étaient ou ont été victimes du cancer du sein de ces femmes dont le monde s’effondre lors du diagnostic ; de ces femmes, mères ou épouses qui se battent pour leur vie et pour la survie de leur foyer de ces femmes qui suivent des traitements lourds aux conséquences onéreuses ; de ces femmes qui guérissent et pour lesquelles la vie ne sera plus jamais comme avant. Le cancer du sein, le plus meurtrier chez les femmes, emporte avec lui chaque année 12 000 mères, sœurs ou amies. J’ai une pensée toute particulière pour elles et pour leur entourage. Aider et soutenir les malades physiquement, psychologiquement et financièrement constitue le cœur de notre système de protection sociale. En commission, nous avons relevé que les prestations médicales et soins de supports, remboursés par l’assurance maladie, n’étaient pas toujours adaptés au quotidien des patientes. Tout d’abord, la répartition inégale de l’offre de soins sur le territoire et les délais d’attente peuvent avoir des conséquences significatives sur les traitements. À titre d’exemple, le coût d’une chirurgie reconstructrice varie grandement et peut dissuader certaines femmes d’y recourir. Cette situation n’est pas acceptable. C’est la raison pour laquelle la commission a adopté l’amendement de la rapporteure, à l’article 1, visant à plafonner les dépassements d’honoraires. Puis, dans le but de réduire le reste à charge pour les patientes, l’article 1 prévoit une prise en charge intégrale de l’ensemble des soins et dispositifs prescrits dans le cadre d’un cancer du sein, ce qui inclut notamment les soins de support, les prothèses capillaires et le renouvellement des prothèses mammaires. Il y a un enjeu indéniable autour de la prise en charge des malades et de l’accompagnement des femmes dans cette épreuve. Cependant, il convient d’apporter quelques nuances en ce qui concerne la prise en charge intégrale des soins jugés spécifiques au cancer du sein, comme ceux qui sont liés à une mammectomie ou à une tumorectomie, et des soins communs dispensés aux patients atteints d’autres formes de cancer. En prévoyant une prise en charge intégrale des prothèses capillaires uniquement pour les assurés atteints d’un cancer du sein et en excluant l’ensemble des autres assurés confrontés à une alopécie consécutive à une chimiothérapie, non seulement nous serions à l’origine d’une inégalité contraire aux principes fondamentaux de notre Constitution,

Cela concerne, par exemple, la prise en charge intégrale des actes de tatouage médical de l’aréole et du mamelon pour les assurées ayant choisi de ne pas effectuer de reconstruction chirurgicale de cette zone, ou encore le renouvellement des prothèses mammaires. En effet, nous ne pouvons accepter que les femmes concernées subissent la double peine de la maladie et du reste à charge des dispositifs médicaux mal compensés par les complémentaires santé.

Plusieurs raisons l’expliquent, comme le manque de temps ou le caractère désagréable de l’examen. Mais le frein réel ne serait il pas la peur du résultat et de la découverte de la maladie ? Le dépistage pourrait pourtant éviter des traitements lourds, douloureux et coûteux.

proposition de loi ne concerne que la prise en charge des soins liés au traitement du cancer du sein, nous avons bon espoir qu’elle constitue la première étape d’un renforcement général des conditions de prise en charge des malades du cancer dans notre pays. Vous l’aurez compris, nous formulons le vœu que l’amélioration des conditions de prise en charge puisse concerner tous les patients, afin d’éviter toute iniquité entre malades. Je pense notamment au cancer colorectal, qui est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme après le cancer du sein. En 2023, toutes populations confondues, presque 50 000 nouveaux cas de cancers du côlon ou du rectum ont été diagnostiqués, et 17 117 personnes en sont décédées. La parole

durant tout le mois d’octobre, nous avons porté le ruban rose, marché, couru, nagé, assisté à des conférences, vendu ou acheté des fleurs, des gâteaux… Et tant d’autres initiatives encore ont mobilisé des dizaines de milliers de nos concitoyens ! Je voudrais commencer par remercier chaleureusement tous ceux – et le plus souvent toutes celles – qui, de la plus grande ville au plus petit village, déploient des trésors d’imagination et d’énergie pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, recueillir des fonds et apporter de la solidarité aux malades. Merci pour eux et pour elles.

On pense souvent que le régime des ALD, qui prend en charge, entre autres, les malades d’un cancer, consiste en un remboursement à 100 %.

qui ont doublé l’an dernier et dont le Gouvernement ne cesse de nous dire que leur évolution n’affecterait pas les malades en ALD, le plafonnement à 50 euros peut conduire à un reste à charge annuel de 100 euros. De nombreuses malades disent subir une double peine : la maladie et son coût financier.

sont à méditer, alors que s’engage le débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et alors que le Gouvernement, madame la ministre, envisage de réduire la part remboursée aux patients par la sécurité sociale sur les consultations médicales

un rapport avait déjà montré que le reste à charge moyen pour une reconstruction mammaire était de 1 391 euros. C’est sans doute bien plus encore aujourd’hui, surtout lorsque les dépassements d’honoraires en lien avec une intervention chirurgicale après une mastectomie peuvent atteindre jusqu’à 10 000 euros. Il n’est pas acceptable qu’une personne qui a combattu la maladie et se trouve enfin sur le chemin de la rémission renonce à une telle intervention, faute de moyens, si elle en éprouve le besoin. Ce problème avait d’ailleurs été soulevé par notre collègue Catherine Deroche, dont la proposition de loi visant à fournir une information aux patientes sur la reconstruction mammaire en cas de mastectomie avait montré que les dépassements d’honoraires constituaient le premier poste de reste à charge pour les femmes.

en un mois, une femme menstruée a dû dépenser de 10 à 15 euros pour l’achat de serviettes, de tampons ou encore d’antidouleurs. Cette même femme, si elle est sous contraception, devra dépenser entre 1,88 et 14 euros par mois pour une plaquette de pilules contraceptives. Ajoutons qu’elle risque d’être davantage confrontée à la pauvreté, avec une carrière plus hachée et plus précaire que ses homologues masculins. Petite remarque : la recherche sur sa santé sera, avec constance, sous financée, et ses particularités bien peu prises en considération en comparaison des affections dont les dont les hommes sont atteints. Cette même femme aura une chance sur huit d’être touchée par le cancer du sein, ce qui entraînera pour elle, en moyenne, 1 300 à 2 500 euros de dépenses supplémentaires dans l’année.

Exemption du reste à charge des forfaits et franchises, prise en charge intégrale des soins et dispositifs prescrits, des prothèses capillaires ou encore des prothèses mammaires : cette proposition de loi, qui sera, je l’espère, votée par les deux chambres en première lecture, crée un précédent essentiel pour les femmes, leur santé et leur situation économique, mais aussi

des femmes atteintes d’un cancer du sein. Plus généralement, quand on voit le Gouvernement s’interroger sur la baisse des remboursements aux personnes en ALD, cette proposition de loi doit nous éclairer et nous permettre de revenir dans le bon sens. Nous comptons sur vous, madame la ministre. Toutefois, même si cette proposition de loi est essentielle pour les femmes atteintes du cancer du sein, elle ne saurait se substituer à des politiques de prévention primaire. Si Octobre rose est un outil de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation intéressant pour le dépistage et l’accompagnement des femmes atteintes d’un cancer du sein, ce n’est toujours pas une politique de santé publique globale.

environ quatre cancers du sein sur dix seraient attribuables au mode de vie, aux expositions professionnelles et à l’environnement en France métropolitaine, avec en première En effet, 15 % des cancers du sein seraient dus à la consommation d’alcool régulière, même modérée. Quant à la pollution de l’air, elle pourrait être responsable de 1 700 cas de cancer du sein chaque année, d’après une étude de l’Inserm de 2022.

Cette proposition de loi constitue un élément clé pour améliorer les conditions de vie de toutes les patientes et pour éviter les renoncements aux soins. Cependant, pour sauver plus de vies, ce modèle devra

d’avoir inscrit à l’ordre du jour de son espace réservé la proposition de loi visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie. Le cancer touche chaque jour près de 1 200 personnes. Un Français sur vingt est concerné, soit deux fois plus qu’il y a trente ans. Le cancer du sein représente 33 % des diagnostics de cancer dans la population féminine. En 2023, près de 61 000 nouveaux cas ont été détectés, ce qui en fait le cancer le plus fréquent chez les femmes. Oui, le cancer du sein est le cancer des femmes, même si 1 % des diagnostics concernent les hommes. L’an dernier, la Caisse nationale de l’assurance maladie recensait plus de 700 000 femmes vivant avec cette maladie. Parmi elles, beaucoup expriment la crainte de ne pouvoir assumer les dépenses non prises en charge, dont le niveau est variable, mais qui s’élèvent à plusieurs centaines d’euros, voire bien davantage. La charge financière moyenne consécutive à un cancer du sein serait comprise entre 1 300 et 2 500 euros. L’attente est donc immense pour venir à bout de cette injustice, qui est d’ailleurs en totale contradiction avec le statut protecteur des ALD. En pratique, En pratique, tous les obstacles financiers du parcours de soins sont loin d’être levés. Plusieurs études ont identifié les principales dépenses à l’origine d’un reste à charge : médicaments peu ou pas remboursés, dépassements d’honoraires, forfaits et franchises, frais de transport, soins de support, cette dernière appellation englobant des produits tels que des crèmes, des activités physiques adaptées, des séances d’ostéopathie ou de suivi psychologique, qui sont pourtant indispensables. Ces soins font partie intégrante du parcours de soins et ne sont ni secondaires ni optionnels ; ils apportent même un peu de confort. C’est là un angle mort de notre système de protection sociale. Selon la Ligue nationale contre le cancer, plus de la moitié des femmes de moins de 40 ans atteintes d’un cancer du sein craignent pour leur budget et doivent faire des faire des choix. Ainsi, 15 % des patientes qui renoncent à une reconstruction mammaire le font pour des raisons financières. De même, la prise en charge des prothèses capillaires et perruques repose en partie sur les complémentaires, ce qui entraîne une répercussion financière non négligeable. De telles situations sont d’autant moins acceptables qu’une ALD est souvent synonyme de baisse des revenus. Peu de personnes atteintes d’un cancer parviennent à maintenir leur niveau de vie ; la maladie peut même les faire basculer dans la pauvreté. Toujours selon la Ligue nationale contre le cancer, une personne sur trois perd son emploi dans les deux ans qui suivent le diagnostic. Il nous revient d’intervenir ; la maladie est en elle même suffisamment éprouvante.

Malheureusement, tel n’est pas systématiquement le cas dans les autres établissements de santé, ce qui est source de grandes inégalités territoriales. Comment peut on accepter que des femmes malades se privent de soins nécessaires pour des motifs financiers ? En ce mois d’Octobre rose, je tiens à dire aux 700 000 femmes atteintes d’un cancer du sein : nous sommes à vos côtés, nous vous soutenons ! Nous voterons bien évidemment pour le texte dont nous sommes saisis aujourd’hui. Cela permettra d’avancer sur la question de la prise en charge du cancer du sein. C’est un premier pas. Mais nous serons aussi d’une extrême vigilance lors du prochain examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. À nos yeux, les efforts de réduction des coûts doivent non pas se faire au détriment des personnes malades, mais être axés sur de meilleures politiques de prévention.

C’est la double peine, et nous ne pouvons l’accepter.

Il est aujourd’hui très rare de ne pas être ou de ne pas avoir été concerné plus ou moins directement par ce type de cancer. Je parlerai beaucoup des femmes dans mon intervention, car elles sont très majoritaires parmi les victimes du cancer du sein,

mais on ne le répétera jamais assez : le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. C’est aussi le type de cancer le plus fréquent en Europe et dans de nombreux pays. Chaque année en France, plus de 60 000 nouveaux cas sont diagnostiqués et l’on sait que 20 000 d’entre eux pourraient être évités. Sur ce point, la période 2022 2023 est malheureusement marquée par une légère diminution du dépistage par rapport à la période précédente. le savons, l’une des principales causes du non recours au dépistage est la crainte de la maladie. Il est parfois plus facile pour certaines de rester dans l’ignorance que d’affronter la peur d’un diagnostic redoutable. Et c’est sur cela que la prévention devrait, selon moi, être axée, sachant que 90 % des femmes traitées à temps d’un cancer du sein en guérissent. Il faut donc absolument parvenir à ancrer dans les mentalités qu’il n’y a pas à redouter un dépistage en ce qu’il y a peu à craindre si la maladie est détectée suffisamment tôt. Malheureusement, pour beaucoup de femmes, les difficultés à bénéficier d’un diagnostic précoce résultent non pas d’un manque d’information ou de sensibilisation à la prévention, mais des difficultés d’accès aux soins dans leur territoire. Les moins chanceuses doivent alors entamer une lutte contre une maladie qui leur coûte beaucoup : physiquement, psychologiquement, socialement, professionnellement et aussi financièrement. Pourtant, sur ce dernier aspect, on ne peut pas dire que rien ne soit fait par notre système de protection sociale. Le cancer du sein est reconnu comme une affection de longue durée, régime permettant une prise en charge plus avantageuse des soins pour le patient, notamment au travers de l’absence de ticket modérateur.

Il reste également les nombreux soins dits de support, mais ô combien nécessaires, et dont le texte suggère la prise en charge intégrale. Par ailleurs, dans la plupart des cas, le cancer n’est pas une maladie invisible. Même si c’est loin d’être l’unique signe du traitement de cette affection, on pense en premier lieu à la perte des cheveux, des cils et des sourcils. Sur ce point, je souhaite rappeler l’aberration que constitue la prise en charge actuelle d’une prothèse capillaire : elle devient nulle si le prix d’achat dépasse les 700 euros, ce qui est justement le cas de la plupart des prothèses de qualité acceptable.

Le débat arrive au bon moment. En cette période d’Octobre rose, de nombreuses actions sont menées. Je remercie toutes les associations et structures en lien avec cette opération de sensibilisation. Il est impossible de ne pas soutenir l’esprit de la présente proposition de loi, qui tente d’adoucir, autant que cela soit possible, le rude combat que doivent mener les personnes atteintes d’un cancer du sein. La parole

Ces éléments statistiques objectifs justifient effectivement que l’on s’interroge sur une meilleure prise en charge des soins liés au traitement du cancer du sein. Comme l’a souligné notre collègue rapporteure, le cancer du sein, considéré comme une ALD, bénéficie de ce fait d’une prise en charge intégrale des frais de santé liés à l’affection à l’affection : chimiothérapie, radiothérapie, mastectomie, chirurgie reconstructrice, pose d’implants et achat de la plupart des prothèses externes. Cette énumération témoigne de l’effort substantiel réalisé au titre de la solidarité nationale. substantiel, il est insuffisant, puisqu’il ne permet pas de financer l’intégralité des dépenses occasionnées par la maladie. C’est vrai, mais je pose la question : de quelles dépenses parlons nous ? S’agit il de dépenses devant relever de l’assurance maladie ?

Permettez moi de rappeler que, depuis décembre 2020, les soins oncologiques de support font partie intégrante du parcours de soins des patients atteints du cancer. Ils sont remboursés par l’assurance maladie. Bien entendu, leur montant est plafonné et, sans doute, limité. ces soins contribuent à une prise en charge globale du patient. Mes chers collègues, vous le savez comme moi, les choix sanitaires sont opérés dans un système qui doit prendre en considération les ressources disponibles.

Je peux partager votre souhait d’offrir aux patientes une prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein. Mais je rappelle que nous avons deux types de financeurs en France l’assurance maladie obligatoire (AMO) et l’assurance maladie complémentaire (AMC). Or je regrette que la proposition de loi n’évoque à aucun moment la contribution financière de ces complémentaires santé dans un domaine qui me semble ressortir de leurs attributions. Une autre dimension fait largement défaut dans le texte : l’absence de référence au développement des dispositifs de prévention et à leur mise en œuvre effective. La La prévention est l’alpha et l’oméga de toute politique de santé. Nous disposons désormais, pour les radiographies des seins, de logiciels d’intelligence artificielle, qui rendent possibles les diagnostics prédictifs. Dans une récente loi de bioéthique,

Ces nouvelles technologies et ces innovations doivent être développées et mises au service de la lutte contre le cancer du sein… et des autres cancers. À côté de la prévention, il y a la sensibilisation – vous en avez parlé, madame la rapporteure. De ce point de vue, Octobre rose est une réelle réussite, car institutions, associations et particuliers se sont approprié le message et le promeuvent souvent dans une approche festive. radiologues (FNMR) : « Octobre rose est bien plus qu’une campagne de sensibilisation. […] En mobilisant la société dans son ensemble, Octobre rose offre un message d’espoir et de solidarité pour un avenir où le cancer du sein n’est plus une menace pour la santé des femmes. »

Derrière cette douce couleur, associée au bonheur et à l’optimisme, se cache une réalité tragique : chaque année, 60 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés en France, et 12 000 femmes en meurent.

rendre tout d’abord hommage aux soignants, à l’engagement des collectivités, mais aussi au tissu associatif et à ses bénévoles. Je pense à la Ligue contre le cancer et à toutes les associations qui œuvrent dans nos départements respectifs pour le bien être des patientes et qui récoltent des dons des dons en faveur de la recherche. En tant que rapporteure pour avis des crédits de la recherche, je veux souligner que nos chercheurs ont impérativement besoin de davantage de moyens pour mieux cibler les facteurs de risque. À Antibes Juan les Pins, comme dans de nombreuses communes de France, nous avons couru, pédalé, nagé et même « régaté », grâce à SOS Cancer du sein, pour sensibiliser dépistage. Notre engagement est également symbolisé par ce ruban rose, qui fleurit sur notre poitrine chaque début d’automne pour rappeler l’essentiel : la prévention. Et pourtant, il reste encore tant à faire. En 2023, le taux de participation au dépistage a chuté. Pire, il est en baisse, et ce depuis dix ans.

au rouge : celui de la colère face aux inégalités d’accès aux soins, notamment dans les territoires ruraux. Cette colère, nous devons la comprendre, mais nous devons surtout y répondre. Saluons ainsi les belles initiatives entreprises

du sein. Malgré le dispositif des ALD, les patientes subissent encore des restes à charge particulièrement lourds, constituant ainsi une forme de double peine, qui s’ajoute à la charge émotionnelle, thérapeutique et sanitaire provoquée par la maladie. De plus, la question du remboursement de certaines dépenses liées aux soins de support, par exemple, ou

les microentrepreneurs peuvent perdre leurs revenus lorsqu’on leur diagnostique un cancer. Si je salue les travaux de Mme la rapporteure sur ces diverses thématiques, je tiens néanmoins à attirer votre attention sur une autre question, qui, comme le dépistage, n’a pas été évoquée dans le texte : l’égal accès des patients aux tests moléculaires. Bien qu’améliorant l’efficacité des traitements tout en limitant les effets secondaires, lesdits tests laissent un reste à charge de près de 50 % aux établissements de santé prescripteurs. Si certains arrivent à en assumer le coût, d’autres ne peuvent tout simplement pas les financer, renforçant ainsi le sentiment d’un système de santé à plusieurs vitesses. Là encore, il faudra certainement que le législateur s’empare de la question.

avant la sénatrice, appelle votre attention. Je ne souhaite pas évoquer ma santé. Néanmoins, que je le veuille ou non, je porte la parole de nombreuses femmes touchées par le cancer du sein. Comme une femme sur huit, j’ai traversé cette épreuve. Le mois d’octobre a marqué une mobilisation de nombreux acteurs contre le cancer du sein. Dans le département de l’Oise, dont je suis élue, j’ai pu participer et soutenir de nombreuses actions. J’ai ressenti une véritable adhésion, tous publics et tous âges confondus. Je suis également membre d’un club de femmes atteintes par le cancer du sein, où nous pratiquons l’aviron et participons à des épreuves sportives nationales et internationales. Cette pratique est encouragée et prescrite par le monde médical. La maladie éloigne, isole, fragilise. Aussi, dans ce combat quotidien, il est essentiel de créer du lien, de savoir que l’on n’est pas seule, de bénéficier de l’expérience d’autres femmes. Encourager et être soutenue sont des remèdes indispensables pour faire face aux traitements et à leurs effets secondaires. Les regards et les mentalités évoluent et nous devons continuer à informer pour toujours mieux dépister. Cette maladie touche tout le monde, à tout âge : le malade, mais aussi son entourage, les aidants ainsi que les proches. C’est pourquoi je soutiens la présente proposition de loi visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie. Évidemment, il n’est pas question de prioriser les maladies. Cependant, j’estime que ce texte constitue une avancée en ce qu’il permettra aux femmes concernées de se sentir reconnues et soutenues. Nous savons que le cancer est un frein pour trouver un emploi et recourir à un emprunt. Si nous pouvons soulager les contraintes matérielles des personnes atteintes d’un cancer, nous aurons déjà fait un grand pas pour les aider à guérir. Enfin,

adaptées est en cours de finalisation. Il doit être adopté d’ici à la fin de l’année – le cahier des charges est quasiment terminé – pour,

de Fabien Roussel pointe fort justement le sujet sensible du cancer du sein et son coût financier pour les personnes qui en sont atteintes. Je voudrais pour ma part insister sur un élément concernant les facteurs de risque de développement d’un cancer. Dans son rapport du mois de juin 2023 sur la santé des femmes au travail, la délégation aux droits des femmes du Sénat avait mis en exergue les conséquences du travail de nuit sur le risque de cancer du sein. Selon les études, le risque de cancer du sein augmente de près de 30 % en cas de travail de nuit chez les femmes non ménopausées. Ce risque augmente encore davantage chez les femmes ayant travaillé de nuit plusieurs fois par semaine sur une longue durée. Ainsi, le risque de cancer est deux à trois fois plus élevé pour les femmes qui ont travaillé plus de deux nuits par semaine pendant plus de dix ans. L’exposition croissante des femmes aux horaires atypiques de travail entraîne des conséquences néfastes pour leur qualité de vie, mais aussi pour leur santé. Cette proposition de loi est donc indispensable pour les infirmières, les aides à domicile, les agents d’entretien – j’en oublie certainement, et j’espère qu’elles m’en excuseront seulement des conditions de travail extrêmement difficiles, mais aussi des risques de développer des cancers supérieurs à la moyenne et,, un reste à charge financier particulièrement injuste.

sur cet amendement. À titre personnel, je ne considère pas que cette proposition de loi soit en contradiction avec le principe d’égalité.

par la sécurisation juridique du dispositif afin de nous assurer que les avancées prévues puissent effectivement entrer en vigueur.

Il était donc nécessaire que le Parlement se saisisse du sujet de l’accès aux soins de support, tant sur le plan financier que sur le plan territorial, puisque de nombreuses disparités existent

satisfait. Vous souhaitez que le Gouvernement remette au Parlement un rapport visant à encadrer la pratique du tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo mamelonnaire pour les femmes ayant subi une mastectomie.

en parallèle le tatouage artistique et non médical, dit tridimensionnel. Pour des raisons de sécurité et de qualité des soins, il n’est pas souhaitable d’élargir la prise en charge de cette technique à des structures non habilitées, les tatoueurs qui la pratiquent n’ayant pas reçu de formation médicale. Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre les cancers, l’Institut national du cancer et le ministère de la santé et de la prévention

Cet article ouvre à la négociation conventionnelle le plafonnement des dépassements d’honoraires relatifs à des actes de reconstruction mammaire. Nous souhaitons que de telles négociations aboutissent

et à propos desquels le Sénat n’a de cesse d’intervenir. J’en veux pour preuve le vote, la semaine dernière, dans cet hémicycle, de la proposition de loi organique d’initiative sénatoriale visant à préserver notre service public audiovisuel en réformant son financement. Aussi, je salue la volonté du groupe CRCE K de placer une fois de plus les services publics au cœur de nos débats. Le texte que nous examinons aujourd’hui se distingue des derniers travaux sénatoriaux sur le sujet. Il s’agit de réviser la Constitution pour protéger nos services publics et leurs usagers.

je rappelle que la norme constitutionnelle n’est pas muette à ce sujet. Dès 1946, le préambule de la Constitution a mentionné les services publics, ainsi que le rôle de l’État dans leur mise en œuvre.

En effet, l’inscription de cette charte dans la Constitution pourrait priver les pouvoirs publics de leur capacité à agir pour faire évoluer les services publics. Elle pourrait ainsi aboutir à un regrettable immobilisme de ces derniers.

La définition d’un périmètre strict a fait l’objet de réserves lors de l’examen du texte en commission. Certains des domaines d’intervention du service public définis par la charte ont semblé hasardeux, à l’image notamment du « développement personnel » de la Nation.

L’instauration par la charte d’un devoir de sauvegarde des services publics renforcerait par ailleurs la « pétrification » du service public, lequel ne pourrait plus évoluer en fonction de nouveaux enjeux d’intérêt général. la charte impose une modification profonde du mode de gestion des services publics, laquelle ne serait pas sans conséquence sur la libre administration des collectivités territoriales. Elle exige en effet de l’État

plus contraignante encore, la charte restreint drastiquement la possibilité pour les gestionnaires publics de recourir à une délégation de service. Ce mode de gestion étant omniprésent à l’échelle des collectivités territoriales, les élus locaux seraient très certainement les premiers à pâtir d’un tel manque de souplesse dans la gestion des services publics.

risque de complexifier encore le cadre juridique que doivent respecter les gestionnaires publics. La majorité des valeurs introduites par la charte découle pourtant des principes d’égalité, de continuité et de neutralité, que la Constitution protège d’ores et déjà. On peut donc estimer que la norme suprême présente aujourd’hui un équilibre satisfaisant. Elle protège des valeurs fondamentales pour nos services publics tout en laissant au législateur le soin de prendre les mesures nécessaires au déploiement concret de ces principes constitutionnels.

dans les premières heures de la construction européenne quant à la préservation du modèle de service public à la française s’est dissipée, le dialogue des juges et le développement des normes ayant permis la conciliation des exigences des deux ordres juridiques. de ces raisons, la commission a jugé que la constitutionnalisation de cette charte ne serait pas en mesure d’améliorer la situation effective des services publics en France. Elle a notamment estimé que la préservation de ces derniers se concrétisera non pas par le désengagement des pouvoirs publics que pourrait engendrer d’une telle charte, mais, bien au contraire, par la mobilisation du législateur et des élus de terrain en faveur du déploiement fin,

Madame la présidente, madame la présidente de la commission des lois, madame le rapporteur,

C’est l’idée que certains besoins appellent une réponse qui ne peut être tributaire de l’initiative privée. C’est l’idée que ces mêmes besoins doivent, au contraire, être pris en charge, autant que nécessaire, par la collectivité tout entière. Parce qu’ils sont essentiels, parce qu’ils sont à la fois la garantie du vivre ensemble et un levier pour mettre en place des politiques publiques, ou parce qu’ils ne peuvent pas ou ne doivent pas dépendre du jeu de l’économie de marché, c’est à la collectivité publique de veiller à leur prise en charge. En France, la notion de service public s’est construite concomitamment – ce n’est bien sûr pas le fruit du hasard – à la conception de l’État moderne. Autrefois défini par ses prérogatives de puissance publique et, selon la conception wébérienne, par son monopole de l’usage légitime de la force, l’État s’est construit au XX siècle comme le garant d’un compromis social qui garantit à tous l’accès à certains services de base : les services publics.

s’agit, avant tout, d’un principe révélant le rôle fondamental que jouent certaines activités pour la cohésion de notre société. En vérité, les services publics sont porteurs de différentes incarnations, selon que l’on se situe du point de vue de l’usager, des agents, des opérateurs économiques, du juriste ou de l’autorité politique. L’éminent professeur de droit public Marcel Waline jugeait ainsi avec humour qu’« il est plus facile de récupérer le mercure échappé d’un vieux baromètre que de saisir la notion de service public La doctrine universitaire s’est bien essayée à trouver une définition du service public. Celle qui est la plus communément admise est attribuée à Gaston Jèze. Selon lui, les services publics sont « les besoins d’intérêt général que les gouvernants, dans un pays donné, à une époque donnée, ont décidé de satisfaire par le procédé du service public ». Dans cette définition, l’intention des gouvernants est déterminante : c’est elle que les critères jurisprudentiels chercheront à identifier. Devant le Conseil d’État, Corneille, commissaire du gouvernement, concluait d’ailleurs : « La notion de service public est une notion en quelque sorte subjective ; elle dépend, pour la plus grande part, de l’intention de l’autorité chargée d’organiser le service. C’est donc une notion révélant le point d’équilibre de notre cohésion sociale, qui varie dans l’espace et dans le temps et structure les choix collectifs. Certains de ces services publics sont aisément identifiables. Ils sont consacrés par nos textes constitutionnels depuis la Révolution de 1789 et constituent l’identité même de notre République. Il en est ainsi de l’éducation : de « l’instruction publique » du constituant de 1791 à « l’enseignement public gratuit et laïc » du préambule de la Constitution de 1946.

de la sécurité sociale posés par le constituant en 1946. La majorité des services publics apparaissent et disparaissent au gré des évolutions de la société et des choix collectifs. Ils ne sont alors pas consacrés par la Constitution, mais ressortissent au pouvoir législatif ou réglementaire. Deux constantes caractérisent cependant le service public dans sa longue histoire : en premier lieu, une expansion continue de son périmètre ; en second lieu, une évolution, voire une reconfiguration de son régime juridique, avec l’essor des modes de gestion privée du service public. Aujourd’hui, les services publics sont confrontés à de nouveaux défis et porteurs d’une formidable capacité de projection de notre société. Identifiés par le Conseil d’État dans son rapport public pour l’année 2022, intitulé, ils requièrent une plus grande ils requièrent une plus grande proximité de l’action publique, ainsi que du pragmatisme et de la confiance. Eu égard à son histoire et à ses enjeux, est il bien opportun d’ériger le service public au rang constitutionnel ? Par ailleurs, les modalités choisies sont elles adaptées ? Je ne le pense pas. D’abord, la notion de service public, aussi essentielle soit elle à l’organisation de notre vie en société, n’a pas sa place dans la Constitution. Ensuite, la charte qui est proposée déstabilisera, à plusieurs égards, l’organisation et le fonctionnement actuels de nos services publics. mes yeux, il n’est pas opportun d’ériger au rang constitutionnel une définition du service public. Aujourd’hui, le service public recouvre les activités identifiées comme telles par le législateur et le juge administratif, selon une jurisprudence bien établie. Celle ci permet de ne pas figer la notion, mais, au contraire, de l’adapter au mouvement constant dont les services publics sont l’objet, pour répondre aux attentes de la société. La jurisprudence du Conseil d’État a défini le service public de manière casuistique, en recherchant toujours l’intention du législateur ou du pouvoir réglementaire, qu’elle soit expresse ou implicite. Procédant à une systématisation de sa jurisprudence, le Conseil d’État a finalement dégagé trois critères d’identification d’une activité de service public. Il s’est d’abord attaché à vérifier le caractère d’intérêt général de l’activité, par nature évolutif et fortement lié à un contexte historique, politique, économique ou social donné. Il a ensuite examiné son lien avec la puissance publique, toute activité de service public étant sinon assurée par l’administration, du moins exercée sous son contrôle. Il a enfin recherché, dans certains cas spécifiques, l’existence de prérogatives exorbitantes du droit commun dont le gestionnaire disposerait pour assurer le fonctionnement de l’activité. Cette approche jurisprudentielle a permis d’éviter deux écueils : une approche trop restrictive du champ des services publics, cantonnés aux seuls services publics régaliens ou traditionnels ; à l’inverse, une approche trop extensive englobant toutes les activités d’intérêt général. Le critère de l’intérêt général a permis d’adopter une approche casuistique et souple du champ des services publics. Quelques exemples célèbres le démontrent. En 1916, le Conseil d’État estimait que le théâtre n’était pas une activité d’intérêt général. au gré des évolutions de la société, et selon certaines circonstances de temps et de lieu, cette même activité a pu recevoir la qualification d’activité d’intérêt général. De même, en matière économique, l’intervention des personnes publiques s’est progressivement affirmée, non d’un bloc, mais avec nuance, afin de respecter le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Le critère de l’intérêt général ne suffit pas à saisir la notion de service public. Le critère organique de la maîtrise de la puissance publique et sa manifestation concrète, le cas échéant prolongée par l’octroi de prérogatives de puissance publique, sont apparus comme indispensables pour encadrer le champ du service public, qui est avant tout une activité pensée et organisée comme telle par les pouvoirs publics. C’est cette intention que recherche le juge administratif dans le silence des textes, à l’aide des critères que je viens d’évoquer. À cette conception souple et casuistique, faisant du service public une notion relative et contingente, la présente proposition de loi constitutionnelle prévoit de substituer une définition unique au plus haut niveau de la hiérarchie des normes.

en droit interne devant toutes les juridictions. pour tous les principes d’organisation et de fonctionnement qu’elle énonce. Ce faisant, elle romprait avec l’état du droit à deux égards. elle élèverait au rang constitutionnel la notion de service public, qui est aujourd’hui une notion le plus souvent de niveau législatif, voire réglementaire. D’autre part, elle graverait dans le droit positif une définition qui, jusqu’à présent, n’existait qu’au travers de critères d’identification élaborés par la jurisprudence. L’opportunité d’un tel rehaussement me paraît discutable. En effet, l’inscription de cette charte dans la Constitution figerait la définition du service public, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Elle conduirait ensuite le Conseil constitutionnel à encadrer l’action du législateur dans un domaine où le choix politique est primordial. En effet, c’est à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il appartient de déterminer, avec vos collègues députés, ce que doit être le champ de l’action publique d’aujourd’hui et de demain. C’est à la loi, que vous vous employez à construire ici, de fixer les règles de fonctionnement du service public et de répondre à l’ensemble des questions que pose aujourd’hui le service public : quel service rendu à l’usager ? Quelles exigences pour l’administration ? Quelles garanties pour le public ? Demain, avec une Charte des services publics, c’est au juge constitutionnel qu’il appartiendrait de déterminer si la loi apporte à ces questions des réponses conformes aux principes qu’elle énonce et à la définition du service public qu’elle grave.

d’abord parce que la définition retenue me semble à la fois imprécise et extensive. Selon le préambule de cette charte, « toute activité qui concerne le développement social, culturel, éducatif, économique et personnel de la société tout entière a vocation à constituer un service public » et l’article 1 dispose que « les services publics concernent les activités indispensables à la réalisation et au développement de la cohésion sociale », sans que l’on sache comment ces deux définitions s’articulent. C’est donc une conception essentialiste du service public, indépendante des circonstances locales et des besoins de la population, que cette charte propose. Le droit raisonnerait non plus en termes de besoin local ou national, de circonstances de temps et de lieu, mais par catégories d’activités. Cela constituerait une rupture majeure avec la conception française du service public. De cette définition, on constate également que le critère organique a disparu. les activités dites de service public seraient non plus seulement celles qui sont assumées ou organisées par les pouvoirs publics, mais toute activité entrant par son objet dans le champ défini. Cela me semble bien sûr inconcevable, surtout si l’on se réfère à une définition aussi accueillante que celle qui est proposée.

incompatibles avec l’organisation actuelle des services publics. En particulier, elle revient de manière radicale sur la possibilité de recourir aux personnes privées pour l’exécution du service public, sauf « nécessité impérative motivée ». Cette disposition est contraire à l’état du droit,

à l’organisation de certains services publics historiques. Je pense bien sûr à la sécurité sociale qui, faut il le rappeler, est gérée à l’échelon local par des organismes et des personnels de droit privé.

la jurisprudence administrative, pleine de sagesse, concilie depuis toujours le principe de continuité à celui de mutabilité des services publics. Cette impression est renforcée à la lecture de l’article 6, qui fait obligation aux gouvernants de « prévenir et de limiter les atteintes aux services publics, qu’ils soient administratifs ou industriels et commerciaux », ou de l’article 7, qui institue un droit de participation des usagers et des agents. De manière générale, il me semble essentiel que le législateur conserve toute latitude pour définir le périmètre des services publics, ainsi que l’étendue et les modalités du service rendu aux usagers. En effet, ces questions touchent au cœur des prérogatives du Parlement : prévoir les principes d’organisation des services publics, déterminer les droits des usagers et définir les orientations budgétaires qui en découlent. Vouloir contraindre les choix exercés en la matière par un texte constitutionnel est une idée contre productive, voire périlleuse. Aujourd’hui, les services publics de notre pays sont confrontés à de nouveaux défis. Plus que jamais, ils sont à la fois plébiscités et critiqués. Leur coût, leur efficacité, leur proximité et leur accessibilité sont autant de questions qui se posent de manière très concrète, service par service, et appellent des réponses pragmatiques. Le temps n’est pas venu de chercher à enrichir notre bloc de constitutionnalité par cette déclaration de principes qui, me semble t il, n’aurait d’autre effet que de venir contrarier la liberté d’action future. Je tiens toutefois à saluer l’ambitieux travail accompli par les rédacteurs de cette proposition de loi constitutionnelle, manifestement inspirés par une haute idée

à l’idée du service public et le souci que nous partageons tous de les faire vivre et de les préserver qui m’amène, mesdames, messieurs les sénateurs, à exprimer l’avis défavorable du Gouvernement sur cette proposition de loi constitutionnelle. La parole est à M.

l’apparition du service public en France est d’abord issue d’un constat dressé en 1871 par le tribunal des conflits : les droits de l’État dans l’exercice d’une activité profitable à tous ne peuvent être les mêmes que ceux des personnes privées. En écho à cette interprétation, le préambule de la Constitution de 1946 mentionne le champ des services publics nationaux : la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs, l’instruction, la formation professionnelle et la culture. publics ne sont pas figés, ils évoluent au gré des besoins du temps et de la société. Pour ma part, je suis attaché à la définition qu’en donne le grand Jaurès : « Le service public est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas.

Ciment de notre solidarité, ferment de notre société et serment républicain, le service public matérialise très concrètement notre ambition collective à vivre ensemble.

Ces décisions, bien souvent verticales, sont vécues comme un arrachement et marquent le déclin irrémédiable d’un État qui se défait. J’ai l’habitude de dire que nos services publics sont l’eau et le sang de l’édifice républicain. Dans une société fracturée, mondialisée, au sein d’un ensemble bringuebalant, le service public est un phare qui nous astreint à tracer la meilleure des voies menant à l’épanouissement de tous et à dresser un rempart contre le fanatisme et l’ignorance.

Le critère du service public est autant l’intérêt général que la solidarité sociale. C’est la mise en commun des richesses d’une nation au profit de chaque individu. C’est l’outil le plus efficace de redistribution et de justice. La dimension territoriale de cette justice est incontournable, mais la réduction des ressources pilotables des collectivités a grandement amputé les marges de manœuvre des élus de proximité.

Cette initiative parlementaire nous offre un débat toujours utile sur les services publics français. Je dis « français » et non « en France », car nos services publics ne s’arrêtent pas à nos frontières. Pour les Français de l’étranger, les services publics sont une manifestation tangible du « faire nation » ; c’est d’autant plus essentiel que ceux ci ne vivent pas sur le territoire de la République. Les services diplomatiques et consulaires sont ce morceau de France qui rattachent à la patrie, ce lien indéfectible qui résiste à la distance.

C’est une charte qui fixe des objectifs sans figer dans le marbre les moyens pour les atteindre. Un texte de cette nature aurait été, à mon avis, plus opportun. Je reviens rapidement sur les arguments plus techniques avancés par Mme le rapporteur, que le groupe

et ce qu’elle représente pour nos 3 millions de compatriotes qui vivent à l’étranger. Les Français de l’étranger sont un laboratoire de modernisation de nos services publics. Ils sont les pionniers de dématérialisations innovantes qui peuvent être pertinentes pour tous les Français. Par exemple, ils ont été les premiers à expérimenter le vote par internet dès 2003, avec un succès certain : lors des élections législatives de 2024, le vote par internet a représenté plus de 75 % des suffrages au premier tour, dépassant les 90 % dans certaines circonscriptions.

Alors que les prises de rendez vous étaient presque devenues impossibles au sortir de la pandémie de covid 19, il est aujourd’hui plus rapide de refaire un passeport dans certains consulats que dans une mairie française ! C’est remarquable et j’adresse mes sincères remerciements à toute l’administration consulaire. Toutefois, ces innovations utiles et nécessaires restent un défi : la fracture numérique frappe nos compatriotes autant à l’étranger que dans l’Hexagone

pas de répondre à une demande croissante, la situation est intenable pour les agents consulaires. Nous serons donc vigilants à ce que la nécessaire prudence budgétaire ne conduise pas à oublier notre service public à l’étranger.

Gageons que nous serons nombreux à défendre, amendement par amendement, l’importance du service public au cours des prochaines semaines. Le groupe Union Centriste ne votera pas cette proposition de loi constitutionnelle. La parole

ans. Un tiers des bureaux de poste a disparu depuis 2010. Quelque 1 200 fermetures de trésorerie et de centre des finances publiques sont

le service public était l’un des éléments qui nous rendaient fiers : la force de l’hôpital public tel qu’il est conçu en France ou celle de la sécurité sociale, qui suscitait chez beaucoup

Sous couvert de simplification, de dématérialisation, d’externalisation et d’optimisation des procédures, nous faisons aujourd’hui les frais de ces politiques d’inspiration néolibérale et des coupes budgétaires qui les accompagnent. Si les grands débats autour de

Il en va de même de l’accueil dans les préfectures. Dans l’immense majorité des cas, il est désormais impossible de pousser la porte d’une préfecture sans avoir préalablement pris un rendez vous en ligne, par exemple pour demander le renouvellement d’un titre de séjour. De telles règles apparaissent comme draconiennes pour certaines personnes et font obstacle, entre autres, à des régularisations. C’est pourquoi nous avons toujours soutenu et continuerons à défendre le droit à un accueil physique dans les services publics. Je souhaite que le Sénat ait prochainement l’occasion de se saisir de cette question primordiale.

l’inscription d’une charte des services publics dans la Constitution présenterait l’avantage de donner aux juridictions constitutionnelles et administratives de nouveaux fondements plus aisément mobilisables pour les protéger. Celles ci pourraient dès lors intervenir pour prévenir la suppression illicite de services publics et garantir leur fonctionnement équitable, notamment en matière d’égalité d’accès. Toutefois, comme l’a fait remarquer la commission, cette charte, telle qu’elle est proposée par le groupe CRCE K, présente quelques imprécisions juridiques qui en affaiblissent malheureusement la portée. Ce n’est guère surprenant, tant la définition juridique du service public est un exercice périlleux.

Malgré ces difficultés sur lesquelles nous souhaitons alerter, nous partageons pleinement la volonté du groupe CRCE K de renforcer nos services publics. C’est pourquoi le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires soutiendra ce texte.

La République s’est honorée en favorisant la prise en charge des besoins élémentaires de tous, notamment des plus démunis, dans l’objectif de renforcer toujours plus l’égalité, la fraternité, ainsi que la cohésion sociale et territoriale.

D’ailleurs, les présidents François Mitterrand et Jacques Chirac ont successivement évoqué la constitutionnalisation de notre conception française du service public, faisant ainsi écho à l’attachement profond dont celui ci fait l’objet.

garantir l’efficience et la proximité des services publics au plus grand bénéfice de nos concitoyens. Ainsi, plusieurs

que celui ci n’est pas adapté à une entrée dans notre loi fondamentale. Lors des crises sociales de ces dernières années, des « bonnets rouges » aux « gilets jaunes », nous avons souvent entendu sur le terrain des revendications qui peuvent se résumer ainsi : moins d’impôts, plus de services publics ! Cette formule n’est contradictoire qu’en apparence 43 % de la richesse nationale produite chaque année dans notre pays est captée par des prélèvements obligatoires. Dans le même temps, nous ne pouvons que constater la dégradation de nombreux services publics : l’hôpital, bien entendu, mais également la justice, les forces de l’ordre et même la défense. Heureusement, le Parlement a récemment adopté plusieurs lois de programmation mettant un terme à ces dynamiques baissières. Il faudra néanmoins beaucoup de temps pour que celles ci produisent pleinement leurs effets et que nos concitoyens ressentent ces évolutions. Environ la moitié des prélèvements obligatoires est affectée à des transferts sociaux, ces sommes sont donc finalement redistribuées aux Français. Si cela est évidemment bienvenu pour ceux qui en bénéficient, c’est autant d’argent qui ne sera pas investi dans les services publics.

de moyens illimités, il est contraint de faire des choix. Nous sommes convaincus qu’il doit se concentrer d’abord sur les missions qu’il est le seul à pouvoir assurer : les missions régaliennes. Il doit ensuite procéder aux investissements structurants pour notre pays. Le reste doit évidemment être laissé au secteur privé. Sans cela, nous continuerions à subir un État qui en fait trop et qui ne peut donc bien faire. Frédéric Bastiat nous met en garde Les finances publiques ne tarderont pas d’arriver à un complet désarroi. Comment pourrait il en être autrement quand l’État est chargé de fournir tout à tous ? Le peuple sera écrasé d’impôts, on fera emprunt sur emprunt ; après avoir épuisé le présent, on dévorera l’avenir. » Nous devons éviter d’en arriver là.

et que nos services publics font partie du patrimoine commun de tous les Français, qu’il s’agisse de l’éducation, de la santé ou encore de la mobilité.

rurales. S’interroger sur la place des services publics au sein même de notre loi fondamentale est donc une démarche parfaitement louable et une initiative qui ne saurait être balayée d’un revers de main.

en matière d’environnement. La singularité de la Charte de l’environnement tient au fait qu’elle ne modifie en rien le bloc de constitutionnalité, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,

K, vous avez repris la même idée en adossant à la Constitution une nouvelle charte, celle des services publics, qui occupent une place essentielle dans notre République et viennent conforter le patrimoine de ceux de nos compatriotes qui en sont dépourvus. Avant d’aborder plus en détail le contenu même du texte, je reviendrai très brièvement sur l’état actuel du droit. Les grands principes régissant le service public sont, de nos jours, dispersés dans plusieurs textes constitutionnels et législatifs, ainsi

C’est donc essentiellement sur l’abondant travail des juges constitutionnels et administratifs, entamé au début du XX siècle, que repose une bonne partie de l’équilibre du service public en France. L’armature législative initialement assez limitée n’a donc pas constitué un obstacle au développement de la conception française du service public. Tout au contraire, elle lui a assuré une certaine forme de flexibilité et d’adaptabilité qu’une constitutionnalisation précoce aurait sans doute beaucoup plus limitée. C’est sur cette flexibilité que ce texte tend à revenir très largement. Pour autant, nous restons très sceptiques sur le contenu même de cette Il est vrai que certains principes y sont gravés dans le marbre, comme la neutralité, l’égalité, l’adaptabilité, la continuité ou encore l’accessibilité. Cela relève bien évidemment de l’évidence.

Ainsi, la formule selon laquelle « les services publics concernent les activités indispensables à la réalisation et au développement de la cohésion sociale » est, vous en conviendrez, difficile d’application, car beaucoup trop large.

vous rigidifiez le système et vous remettez indirectement en cause la capacité d’action des pouvoirs publics en matière de gestion des services publics. Une telle évolution est susceptible de toucher tout particulièrement l’échelon local, même si je peux en comprendre la philosophie sous jacente : par cette disposition constitutionnelle, vous posez en quelque sorte les limites de la privatisation de grands services publics tels que l’armée, la justice, la police, la monnaie ou les prisons. En d’autres termes, existe t il des limites à la privatisation ? Il est vrai que les efforts déployés par le secteur privé, encouragés parfois par l’Union européenne, pour coloniser le cœur de l’État, ou tout au moins y établir des protectorats, donnent à la question une saveur toute particulière. Pour autant, je vous renvoie à ce que le Conseil constitutionnel a jugé dans quatre décisions rendues à propos de projets de loi de nationalisation et de privatisation de 1986 à 1996 à 1996 : il existe des services publics dont « l’existence et le fonctionnement [peuvent être] exigés par la Constitution ». Ces décisions marquent donc l’ébauche d’une éventuelle nouvelle catégorie de services publics, dont le contenu constituerait une réserve à la compétence du législateur : certains services publics existeraient de par la Constitution, de telle sorte que le législateur ne pourrait ni les amputer

que l’État doit être le garant ultime du fonctionnement et du financement des services publics. Cela ouvrirait incontestablement une brèche dans le principe de libre administration des collectivités territoriales en permettant une forme de tutelle de l’État sur celles ci.

En agrandissant toujours plus le sommet de la pyramide de la hiérarchie des normes, nous courons le risque d’engendrer une forme d’impuissance des niveaux inférieurs, à commencer par celui qui relève du pouvoir législatif, c’est à dire le nôtre.

les uns aux autres et hiérarchisés par l’unique arbitre en la matière : le juge constitutionnel ? Leur solennité s’en trouverait nécessairement dévalorisée.

mais nous craignons fort que le choix de constitutionnaliser les principes fixés dans cette charte n’aboutisse en définitive à un désordre et à une paralysie juridique

La notion de service public dépasse largement la simple organisation d’infrastructures ou de moyens humains. Elle incarne les valeurs et les principes d’égalité, de solidarité et de justice sociale qui sont les piliers de notre République. Avoir accès aux services publics, c’est pouvoir jouir de nombreux droits fondamentaux, tels que le droit à la santé, au logement, à l’éducation ou à l’hébergement d’urgence. Lorsque le service public faillit, c’est la cohésion nationale elle même qui se fragilise.

Nos territoires ultramarins connaissent des réalités géographiques et économiques spécifiques qui appellent des réponses sur mesure pour garantir l’égalité républicaine. de notre territoire, des services accessibles et de qualité sont indispensables, non seulement pour accompagner les Français dans leur vie quotidienne, mais également pour bâtir une République plus solidaire. Dans ce contexte, la constitution du réseau France Services offre un exemple concret de solution rapprochant le service public des Français. Les 2 840 espaces recensés répondent aux besoins des zones rurales et périurbaines, redonnant vie à des territoires parfois dépourvus d’infrastructures adaptées et offrant un accompagnement de proximité. La Cour des comptes en a récemment dressé un bilan plus que positif : le nombre de demandes traitées est passé de plus de 1 million en 2020 à près de 9 millions en 2023, preuve que l’État est capable d’innover pour mieux servir nos concitoyens. En intégrant une charte des services publics au bloc de constitutionnalité, la proposition de loi constitutionnelle que nous examinons aujourd’hui entend mieux préserver et assurer un fonctionnement pérenne de l’ensemble des services publics. Je comprends l’intention des auteurs de ce texte et salue leur travail pour soumettre ce sujet au débat. Cependant, le véhicule législatif et la rédaction choisis ne nous semblent pas servir leurs objectifs. Ils risquent au contraire de perturber significativement l’organisation des services publics, déjà bien établie, et reposant principalement sur la jurisprudence du Conseil d’État. En effet, le champ retenu à l’article 1 de la charte supprime le critère organique inhérent au service public. Il ne permet plus d’identifier l’organisme, public ou privé, chargé de la mission de service public, c’est à dire la personne qui l’assume, que ce critère constitue l’essence même de la construction de notre droit. La définition proposée paraît à la fois trop rigide et trop large, au risque d’accroître de manière incertaine le domaine d’intervention des pouvoirs publics. En ces termes, cela serait de nature à compromettre la gestion efficace des services publics par les collectivités et les pouvoirs publics. De la même manière, ériger une définition des services publics au niveau constitutionnel peut limiter la souplesse de ces derniers et complexifier leur adaptation aux réalités économiques qui évoluent constamment.

en imposant à l’État d’être le garant du fonctionnement pérenne des services publics, l’article 4 expose les collectivités territoriales à un risque de contrôle accru de la part de l’État, mettant en péril le principe de libre administration consacré consacré par l’article 72 de la Constitution. Si l’accès de tous à des services publics de qualité est un objectif naturellement partagé, il est délicat de modifier la Constitution de cette manière, au risque de diluer son caractère fondamental et de l’exposer à des révisions opportunistes.

ce texte ne permet malheureusement pas d’atteindre les objectifs annoncés. C’est pourquoi nous y serons défavorables. La discussion La discussion générale est close. La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi constitutionnelle initiale.

Mes chers collègues, je vous rappelle que, si cet article n’était pas adopté, il n’y aurait plus lieu de voter sur l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle, dans la mesure où les deux articles qui la composent auraient été supprimés. Il n’y aurait donc pas d’explications de vote sur l’ensemble.

Sénat n’a pas adopté. Les deux articles de la proposition de loi constitutionnelle ayant été successivement supprimés par le Sénat, je constate qu’un vote sur l’ensemble n’est pas nécessaire puisqu’il n’y a plus de texte. En conséquence, la proposition de loi constitutionnelle instaurant